alimentaires, rendant le réemploi ou le don impossible, pour une orientation directe vers le recyclage ou la destruction. Il tend à suivre la même logique que les dispositions introduites par la loi Garot sur le gaspillage alimentaire. Quel est l'avis de la commission

lesquels sont tous susceptibles d'être en relation commerciale au sein d'une même chaîne d'approvisionnement. Compte tenu des risques de déséquilibre déjà existants au sein des relations entre distributeurs et fournisseurs, ces derniers craignent que le risque commercial de la gestion des invendus ne se reporte exclusivement sur eux, en particulier dans le cadre des conventions annuelles à venir. Il convient donc de rappeler de façon explicite l'application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, ce qui permettra en outre de se prémunir contre des atteintes aux réseaux de distribution sélective.

Plus tôt dans l'après-midi, on rappelait justement à quel point il était important d'éviter les exceptions ou les restrictions, pour laisser le champ le plus libre possible

n° 40 rectifié . La vente des invendus non alimentaires au personnel de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, moyennant une réduction tarifaire, permet d'offrir une seconde vie aux produits qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus. L'organisation de ce type de vente constitue un débouché naturel de ces invendus qui n'ont pas trouvé d'acquéreur au cours de leur période normale de commercialisation. Les ventes au personnel répondent à un triple objectif écologique, économique et social, cette voie d'écoulement des stocks étant complémentaire des donations effectuées en faveur d'opérateurs du don à à des personnes en situation de précarité. Le droit actuel en matière de vente au personnel repose sur une ancienne position administrative peu compatible avec les enjeux sociaux, économiques et écologiques en présence.

préférentiel à leur personnel, les privant d'une solution d'écoulement des stocks invendus. Cet amendement vise donc à assouplir le régime social de ces ventes à tarif préférentiel afin de faciliter l'écoulement des invendus au sein du personnel de l'entreprise concernée. Afin de lutter efficacement contre les invendus non alimentaires,

est l'avis de la commission ? Actuellement, les produits invendus qui sont remis gratuitement par les entreprises à leurs salariés ou qui leur sont vendus à un prix ne dépassant pas 30 % de leur prix de vente sont considérés comme des avantages en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG. Ces amendements identiques visent à exonérer de CSG ces produits s'ils sont remis gratuitement aux salariés ou vendus à des conditions tarifaires préférentielles, dans la limite du seuil de revente à perte. Ils tendent à favoriser le don à la vente des produits invendus aux salariés qui ont participé à leur conception et ont donc une dimension à la fois environnementale et sociale.

La loi Garot, promulguée en février 2016, vise à lutter contre ce gaspillage, et la loi Égalim a étendu l'obligation

de voir leur responsabilité engagée en cas d'incident. L'Ademe pointe ce sujet de l'éducation et de la formation des employés, en soulignant que des efforts devraient avoir lieu à chaque étape : production, transformation, distribution et consommation.

par exemple des modules d'e-learning Certaines associations le font déjà et indiquent que le management des grandes et moyennes surfaces a beaucoup évolué grâce à cela. En revanche, obliger tous les personnels des grandes surfaces à se former sur le sujet paraît disproportionné.

Ce texte prévoit déjà que les distributeurs mettent en place un plan de formation des personnels chargés de la réalisation des dons.

pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur. Or ce délai d'au moins deux ans à compter de l'entrée en vigueur prévisionnelle de la présente loi semble excessif au vu de la nécessité d'interdire le plus rapidement possible cette pratique qui s'oppose à la nécessaire lutte contre le gaspillage. Il n'y a pas de honte à être un bon élève en matière de vise donc à ramener ce délai au 1 janvier 2021, ce qui semble plus acceptable. Les entreprises auront un an pour comprendre qu'elles doivent arrêter de détruire du neuf et de surproduire, ce qui semble amplement suffisant.

en particulier à celles qui sont assujetties à de nouvelles obligations, le temps de s'y préparer. S'agissant de l'interdiction de la destruction des invendus, les entreprises concernées doivent s'organiser pour définir les modes de traitement les plus adaptés, lorsque la loi aura été promulguée et son aura été promulguée et son décret d'application pris. Par conséquent, il ne nous semble pas souhaitable de modifier les dates d'entrée en vigueur prévues à l'article 5. L'avis de

aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits mis sur le marché, afin de lutter contre le gaspillage. Il ne saurait cependant s'appliquer à des produits qui étaient déjà soumis aux règles de responsabilité élargie du producteur, mais pour lesquels il n'existe pas encore de solution de recyclage pour un produit ou une matière donnée. C'est le cas notamment des chaussures en cuir. Les chaussures appartiennent à la filière relevant de la responsabilité des producteurs textile, linge de maison et chaussures, mise en oeuvre en 2007. Or, à ce jour, et après désassemblage, les chaussures en cuir ne peuvent être totalement recyclées, le traitement du cuir demeurant complexe. Il en va de même pour certains produits d'habillement confectionnés à partir de matières multiples. de matières multiples. Cet amendement vise donc un allongement du délai d'entrée en vigueur de l'article 5, pour permettre à la filière de mettre en oeuvre des solutions adaptées. est l'avis de la commission ? En réalité, l'existence d'une filière REP suppose l'existence d'une filière permettant de gérer la fin de vie du produit. En tout état de cause, une dérogation déjà prévue permet, lorsque le dispositif entre en vigueur, de ne pas assujettir au dispositif les invendus pour lesquels les conditions nécessaires pour réaliser leur réemploi,

pour les produits non soumis au principe de REP. Le texte actuel prévoit un délai courant jusqu'au 31 décembre 2023, soit potentiellement quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi. Une fois de plus, ce délai nous semble excessif et n'encouragera pas les entreprises concernées à changer leurs habitudes dans l'immédiat.

l'amendement n° 119. Par cet amendement, nous souhaitons mettre en lumière et rectifier plusieurs pratiques. Nous voulons tout d'abord lutter contre le gaspillage alimentaire et mettre fin à une injustice que subissent les habitants des outre-mer. Nous voulons qu'un décret fixe les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimales sur les produits alimentaires, afin d'assurer une mise en oeuvre uniforme. Pour certaines catégories de produits, le producteur choisit lui-même la date d'utilisation optimale qu'il place sur ses produits. Le consommateur est tellement conditionné par ces dates qu'il finit par être piégé et ne fait plus appel au bon sens pour savoir si un produit est périmé ou pas. Les producteurs, marques et distributeurs peuvent de leur côté avoir un intérêt commercial à ces inquiétudes, voire les encourager. Les dates de durabilité minimale, ou DDM, sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables sur lesquels elle est inutile, voire trompeuse. La DDM est également trompeuse, car elle laisse croire qu'elle donne une information sur le caractère consommable d'un produit, alors qu'elle indique seulement une date où le produit peut perdre certaines de ses qualités gustatives ou de texture. Les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables après la date indiquée. Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation peuvent varier selon qu'il est commercialisé sur le territoire métropolitain ou ultramarin. Elles sont alors allongées afin d'assurer le temps de sa commercialisation. Il s'agit donc non pas d'un principe de précaution, mais d'une tactique commerciale qui favorise le gaspillage de produits alimentaires- cela représente près de 20 % des dix millions de tonnes gaspillées chaque année. L'encadrement global des différentes dates d'utilisation est fixé au niveau européen. Nous en souhaitons une déclinaison nationale établie, par décret, afin d'assurer une cohérence dans l'apposition de celles-ci par grandes familles de produits. Nous avons adopté en commission une demande de rapport sur les dates d'utilisation des produits alimentaires. Or le sujet est déjà suffisamment documenté pour ne pas le remettre encore une fois à plus tard. Les initiatives existent : le groupe Carrefour a déjà retardé la date de péremption sur près de sur près de cinq cents de ses produits sans en changer la composition ; les producteurs de lait norvégiens ont récemment changé la formulation des dates afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous parlons de 2 millions de tonnes d'aliments qui ont été produites, emballées, transportées, puis jetées.

Nous pensons que la date de durabilité minimale et les dates limites de consommation contribuent au large du gaspillage alimentaire dans notre pays, en incitant le consommateur à jeter des produits qui seraient encore consommables. On trouve dans nos poubelles 10 % de produits alimentaires qui n'ont pas été ouverts. Par ailleurs, sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Les dates sont souvent allongées outre-mer, afin d'assurer leur commercialisation. Nous sommes donc très éloignés d'une mesure de précaution et d'une mesure sanitaire. L'encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d'assurer une cohérence dans la fixation de celle-ci par grandes familles de produits.

une mise en oeuvre uniforme des DLC et DDM sur le territoire national. Deuxièmement, les dates limites de consommation appliquées par les industriels sur leurs produits frais ont connu d'importantes modifications ces dernières années, dans un sens favorable au combat contre le gaspillage alimentaire. Troisièmement, et enfin, il s'agit, comme nous l'avons déjà dit, d'un sujet réglé au Nous avons, en ce sens, complété l'article 5 en commission par un IV prévoyant la remise d'un rapport évaluant l'impact des DLC et des DDM sur le gaspillage alimentaire, rapport qui devra précisément jeter les bases d'une position défendue par la France, afin de faire évoluer la réglementation européenne.

J'ai moi-même, dans une autre fonction, fait voter un texte visant à harmoniser les dates limites de consommation entre l'Hexagone et les outre-mer. Le texte existe

Il vise à prévoir que les acteurs du domaine de la santé peuvent conclure des conventions en vue de céder à des associations à titre gratuit du matériel médical pour le reconditionner. Il convient en effet de favoriser le réemploi du matériel médical. Cette démarche est aujourd'hui rendue possible grâce aux acteurs de l'économie circulaire du domaine de la santé. En obligeant les établissements de santé à prévoir le réemploi de leur matériel médical usagé et en incitant les particuliers à faire réparer ou recycler le leur, nous permettrons une meilleure accessibilité financière de ces biens pour les patients les moins favorisés. Cela permettrait également de réduire les dépenses de la sécurité sociale, tout en créant des emplois dans le domaine de l'économie circulaire. Quel est l'avis de la commission ? L'objectif

: La parole est à Mme Martine Filleul. Parmi les mesures importantes de ce texte figure l'interdiction de la destruction des invendus. C'est une mesure qui est réclamée depuis longtemps par les associations de protection de l'environnement et qui va tout à fait dans le bon sens, ne peut être totalement satisfaisante, car il faut travailler sur l'amont et réfléchir à la manière dont nous produisons pour éviter d'en arriver à de telles situations. telles situations. Il faut donc réfléchir à nos modes de production et aux quantités que nous produisons. La surproduction, ce surplus de marchandises par rapport à la demande des consommateurs, est non seulement inutile, mais elle est en partie responsable de la destruction de la planète. C'est pourquoi l'amendement qui vous est présenté, mes chers collègues, vise à inscrire dans le code de l'environnement le principe de la lutte contre la surproduction, en mobilisant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations.

Dans le cas de la vente en vrac, cela ne pose aucune difficulté. En revanche, dans le cas de la vente à la coupe- boucherie, fromagerie, poissonnerie, boulangerie ... -, des questions se posent. Cette pratique se développe de plus en plus, et des consommateurs demandent à leurs commerçants de les servir dans des contenants- récipients, bocaux ... -qu'ils ont apportés. Certains commerçants se prêtent volontiers à cette pratique. D'autres s'inquiètent légitimement de leur éventuelle responsabilité, si le contenant du consommateur venait à contaminer leurs produits ; du coup, ils refusent de procéder ainsi. Cet amendement a pour objet de fixer un cadre légal à cette pratique, comme l'a d'ailleurs envisagé le Premier ministre en août dernier,

Cet amendement est donc tout simple ; il vise à apporter une sécurité juridique à une pratique vertueuse de nos concitoyens. Il serait vraiment dommage de brider une telle pratique, vertueuse, je le répète, pour cause d'insuffisance du droit. Précisons, pour finir, que ce cadre juridique est en vigueur chez nos- remarquables -voisins belges

Cet amendement tend également à préciser que la vente en vrac d'un produit ne peut être interdite que pour des raisons de santé publique. Il nous semble en effet indispensable de donner un cadre juridique à cette pratique vertueuse qui est très répandue en France. Cette proposition émane d'ailleurs d'une très forte demande du secteur qui pâtit aujourd'hui de l'absence de normes, et il nous semble nécessaire d'entendre cette demande. Je rappelle que la vente

un contenant réutilisable, afin de procéder à ses achats. Cette proposition s'inscrit totalement dans la ligne de la commission visant à réduire les quantités d'emballages.

Pour des raisons relevant souvent de la certification de l'origine, de nombreux cahiers des charges de signes d'identification de la qualité et de l'origine- SIQO -ne prévoient pas la possibilité pour les commerces de détail d'ouvrir les emballages des produits et de les transvaser dans les équipements de vente en vrac. Tel est le cas, par exemple, des cahiers des charges des SIQO suivants : noix de Grenoble, lentilles du Puy, riz de Camargue, vinaigre de Modène. Pour beaucoup de ces produits, la vente en vrac est une évidence- sans surprise, je prendrai l'exemple de la noix de Grenoble. Pourtant, les produits sous SIQO sont recherchés par les consommateurs qui achètent en vrac, la qualité et l'origine constituant des piliers pour une consommation responsable et durable. Cela se vérifie particulièrement pour les produits secs, tels que les pâtes, le riz, les lentilles, les haricots ou les fruits secs. Leur vente en vrac représente ainsi un important débouché pour les SIQO. Il est regrettable qu'il ne soit pas systématiquement tenu compte de cette modalité de vente lors de l'élaboration des cahiers des charges des SIQO, qui doivent comporter une partie sur la vente en vrac et les protocoles à mettre en place par les commerçants pour garantir la qualité et la traçabilité des produits. De tels protocoles existent d'ailleurs déjà dans la plupart des cahiers des charges des produits frais sous SIQO- fromage, charcuterie -qui peuvent être vendus à la coupe, c'est-à-dire non préemballés. Aussi, il convient d'imposer que les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévoient les conditions, dans lesquelles les produits sont vendus en vrac. est l'objet de cet amendement. Le

vente en vrac. En outre, l'amendement n° 221 vise à imposer sans délai une révision de tous les cahiers des charges ; le sous-amendement tend à restreindre cette disposition à ceux qui ne prévoient pas déjà la vente en vrac et à demander aux autres de justifier la non-prise en compte du vrac ou d'engager une révision pour la prévoir sous trois ans.

fait face à des difficultés réglementaires fortes, faute de volonté politique affirmée. Afin de renforcer son attractivité et de s'assurer qu'elle participe clairement au renforcement du pouvoir d'achat des consommatrices et des consommateurs, nous proposons d'agir sur le taux de TVA qui affecte les produits non emballés en libre-service dans les grandes surfaces. Ainsi, nous proposons d'exonérer les produits alimentaires vendus en vrac, aujourd'hui taxés au taux de 5,5 %. Une telle disposition semble juste et souhaitable, lorsque l'on sait que la vente directe des agriculteurs aux consommateurs est également exonérée de TVA. Nous proposons parallèlement de fixer le taux de TVA des produits non alimentaires à 10 % au lieu de 20 %. Il s'agit d'un exemple concret permettant de conjuguer l'exigence d'un renforcement du pouvoir d'achat de nos concitoyens et la nécessaire transition écologique. Il faudra ensuite que le Gouvernement porte cette exigence auprès des instances européennes, afin de la rendre effective. Nous considérons que cette filière fragile doit bénéficier d'un réel soutien des pouvoirs publics et l'outil de la TVA nous semble particulièrement adapté pour ce faire. Nous espérons donc que cet amendement sera adopté. Quel

la TVA. J'entends qu'il y a un monopole des lois de finances, mais je n'en crois rien. À mon sens, nous pourrions dès ce soir décider de baisser la TVA sur les activités de réparation.

Réparer un objet ou un appareil permet de prolonger sa vie et de réduire les déchets à la source. Cependant, le coût des activités de réparation est souvent très proche, voire supérieur au prix du produit neuf, de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe, estime en effet que seuls 44 % des appareils qui tombent en panne sont réparés. En complément d'autres mesures relatives à l'allongement de la durée de vie des produits -amélioration de leur réparabilité, extension des garanties des constructeurs, obligation de produire les pièces de rechange pendant cette durée -, l'une des pistes d'action pour rendre la réparation plus attractive consiste à appliquer un taux de TVA réduit sur les activités de réparation, afin de faire diminuer son coût et inciter le consommateur à utiliser ce service. Le réemploi et la réparation permettent en outre de créer de l'emploi local, bien souvent dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Ces activités doivent être soutenues, notamment avec un taux de TVA réduit sur la vente des produits de seconde main, qui ont transité par une filière de réemploi ou de réparation. Cet amendement vise donc à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparation en le fixant à 5,5 %. Il s'agit d'encourager ce secteur d'avenir, en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille de route économie circulaire du Gouvernement.

il est préférable de réduire ce coût grâce au fonds de réparation abondé par les éco-contributions des éco-organismes, tel que la commission l'a voté, plutôt que par des incitations fiscales pesant sur le budget de l'État. L'amendement

? Nous pensons qu'il est indispensable de passer par les éco-organismes. Il faut nous appuyer sur eux pour développer et structurer l'offre de réparation. Notre principal levier sera de fixer aux éco-organismes des objectifs clairs, mesurables et chiffrés

produits. Enfin, nous voulons que les éco-organismes travaillent de façon plus ciblée et plus efficace à créer des réseaux de réparateurs. Nous pensons que c'est plus ciblé et plus efficace

et une moyenne de 30 kilos annuels par foyer. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable, pour l'environnement, bien évidemment, mais aussi pour la collectivité et pour nos concitoyens.

ont été retoqués au nom de l'article 45 de la Constitution. Pourtant, d'après nous, ils avaient un lien direct avec le texte, puisqu'ils poussent outrageusement et continuellement à la consommation, ce qui constitue une pollution lumineuse, ainsi qu'un gaspillage de ressources et d'énergie. Nous le disons depuis le début de nos travaux, nous devons changer notre modèle de consommation et en nous en donner les moyens.

près de 3 milliards d'euros en 2017, auxquels il faut bien sûr ajouter le coût de collecte et de traitement des déchets pour les collectivités et les citoyens. À ces dépenses s'ajoute encore le coût environnemental de la fabrication de papier, très consommatrice en eau et en énergie : l'impact d'une tonne de papier est estimé à une tonne de CO2. Le dispositif « Stop pub » a permis de diminuer le nombre de prospectus distribués, mais il rencontre aujourd'hui certaines limites. Par souci de clarté, et avec l'ambition de voir enfin diminuer drastiquement la diffusion de publicité papier non adressée, nous vous proposons d'inverser la logique du « Stop pub » en autorisant la distribution de prospectus dans le seul cas où une mention l'y autorisant figure sur la boîte aux lettres. Cette mesure simple serait un signal fort donné à nos concitoyens, qui rejettent pour la plupart ces sollicitations en nombre et qui sont demandeurs d'actes concrets en matière de réduction des déchets.

Ces différents amendements ont pour objet la distribution d'imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres. Ils visent à inverser le principe applicable.L'objectif

sur lequel pèsera la responsabilité -distributeur ou enseigne pour le compte de laquelle la publicité est distribuée. Ensuite, l'inversion du principe peut susciter des inquiétudes d'ordre social, car il stigmatisera celui qui fera le choix d'afficher un logo « Oui à la pub » et il privera certaines populations d'informations auxquelles elles peuvent être attachées. Je pense notamment, pour les connaître dans mon arrondissement, à certaines personnes âgées ou isolées, pour lesquelles cette distribution peut constituer une forme de lien social et qui ne seront sans doute pas les mieux

constatons tous le caractère hyper intrusif et excessif des publicités dans les boîtes aux lettres. Même lorsque vous faites la démarche volontaire d'essayer de l'éviter, cela n'est pas toujours respecté.

je me sens bien dans le groupe RDSE ; je tenais à vous le dire.

Cela étant, je vais prendre le contre-pied de mon collègue François Bonhomme. Je crois que nous sommes dans une société où il faut laisser la liberté et le choix à nos concitoyens, en responsabilité. En tant que maire, j'ai eu l'occasion de travailler sur ces sujets. Nous avions distribué à l'ensemble de nos concitoyens et à tous les foyers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

Cet amendement vise à interdire la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale, lorsque celle-ci n'est pas sollicitée par les consommateurs. Cette nécessité nous semble totalement en phase avec l'objet du présent projet de loi en matière de lutte contre le gaspillage. Selon certains chiffrages, quelque 18 milliards d'imprimés, soit 800 000 tonnes de papier ou 30 kilos par foyer par an, transitent ainsi dans nos boîtes aux lettres. Nous devons mettre un terme à cette source importante de déchets, qui, de plus, participent souvent de méthodes commerciales agressives pouvant s'apparenter à du harcèlement, tant nos boîtes aux lettres peuvent être polluées, dans tous les sens du terme, par ces prospectus. En outre, nous visons les publicités contenant des huiles minérales, qui sont non biodégradables et polluantes.

à M. Joël Bigot. Cette proposition vient faire écho à l'engagement signé en juin 2019, par seize enseignes de la restauration rapide, de faire en sorte que 70 % de leurs restaurants soient en conformité avec la législation en vigueur en matière de tri des déchets d'ici à la fin de l'année 2019. pouvons tous constater, lorsque nous nous rendons dans ce type de restaurant, que la réglementation du tri dit « 5 flux » n'est pas respectée. Ainsi, tous les détritus, emballages, papiers, cartons, plastiques et aliments se retrouvent dans la même poubelle. Cette situation, qui est une aberration écologique, est d'autant plus dérangeante qu'elle n'est pas en conformité avec le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Comme beaucoup, je suis surpris de constater que, au lieu de sanctionner ces enseignes, nous acceptons des engagements finalement peu contraignants. C'est pourquoi nous demandons la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement

Je pense à ce stade, monsieur le sénateur, que les demandes que vous formulez sont satisfaites et je suis tout à fait prête à partager les informations avec vous, parce que je considère qu'elles doivent être du domaine public. Je sollicite

ou encore l'affichage du débit d'absorption spécifique pour les téléphones portables, il nous semble opportun d'informer le consommateur pour lui permettre d'orienter son choix vers des produits plus durables et plus vertueux. Nous voulons, avec cet amendement, rendre obligatoire dans les publicités des informations relatives aux caractéristiques environnementales, à l'indice de réparabilité et aux consignes de tri.

La meilleure manière de limiter la production de déchets est de limiter la consommation de produits neufs, quand il s'agit du remplacement de produits détériorés. Pour passer de la culture du jetable à la culture du durable, il est indispensable de transmettre à l'ensemble de nos concitoyens le réflexe d'essayer de réparer avant de remplacer. À la manière d'autres mentions d'intérêt général, comme celles qui sont relatives à la consommation d'alcool ou de produits gras et sucrés, il est indispensable d'accompagner la publicité d'une mention informative pour faire évoluer les comportements.

Mes chers collègues, le secteur de la construction représente aujourd'hui une part non négligeable de la production de déchets, avec près de 230 millions de tonnes produites chaque année, soit environ 77 % des déchets français uniquement pour le secteur de la démolition. Aujourd'hui, seuls 5 % à 10 % des chantiers réalisent vraiment un diagnostic « déchets », pour de multiples raisons. L'extension du recours au diagnostic, qui est prévue à l'article, va dans le bon sens, mais ne me semble traiter qu'une partie minime du problème. La démolition n'est que l'avant-dernière étape de la vie d'un matériau, avant sa réutilisation ou avant son recyclage. me paraît d'ailleurs nécessaire de souligner l'importance de traiter la question des déchets le plus en amont possible, afin d'être plus exigeant sur la date de construction.

Je sais que ce n'est pas simple, et je prendrai un exemple tout à l'heure, mais cela me paraît important. Nos règles d'urbanisme doivent donc évoluer. On ne peut plus, aujourd'hui, se contenter de bâtiments dont l'avenir se limite à quelques décennies et qui sont ensuite, pour le dire poliment, « déconstruits

l'éco-conditionnalité. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le renforcement du diagnostic « déchets » avant démolition est utile, mais ce n'est en fait qu'une partie du problème. Sur ce sujet, comme sur d'autres, il nous faut assurément élargir le cadre de la réflexion pour prendre en compte le devenir des produits à partir de l'analyse de leur cycle de vie, notamment en l'état actuel des connaissances. En disant cela, je pense notamment, dans les matériaux de construction, aux plaques de fibrociment qui contiennent de l'amiante : à l'époque où elles ont été vendues, elles avaient tous les labels nécessaires, et l'État donnait, bien évidemment, son blanc-seing.

Mme Josiane Costes. D'après l'étude d'impact, le secteur du bâtiment et des travaux publics suscite 228 millions de tonnes de déchets sur les 324 millions de déchets produits en France. Plusieurs mesures proposées par le projet de loi visent à mieux gérer ces déchets, parmi lesquelles l'extension de l'application du diagnostic « déchets » aux opérations de démolition ou de réhabilitation significatives des bâtiments, alors qu'il est actuellement réservé aux opérations lourdes. Afin de rendre effectif ce dispositif, il convient de déterminer par décret une surface minimale de plancher

En effet, ce dernier étend le périmètre du diagnostic « déchets » et précise ses conditions de mise en oeuvre. Il faut dire que les déchets du bâtiment et des travaux publics constituent une problématique forte, puisqu'ils représentent un quart des déchets produits en France. La commission a complété ce dispositif par des éléments sur la traçabilité, qui constitue une forte attente des acteurs de la filière aval et des collectivités territoriales. Les architectes participent à ces exigences en imaginant, en amont, la construction et l'utilisation de matériaux moins producteurs de déchets, participant ainsi à la nécessaire transition écologique. Notamment, à la lumière de leur expérience de chantiers de déconstruction/démolition, les architectes pensent que l'article 6 pourrait être utilement complété en précisant les filières de recyclage existantes dans le diagnostic préalable, en sécurisant la réutilisation des produits et matériaux récupérés compte tenu des enjeux assurantiels existants, et, enfin, en prévoyant les modalités d'élimination ultime des déchets.

et des déchets de la démolition ou de la réhabilitation et à le préciser en incluant l'élimination des déchets qui ne seraient pas recyclables. Un tel encadrement permettrait de sécuriser l'atteinte des objectifs en termes d'économie circulaire, tout comme il garantirait l'assurabilité de la nouvelle mission du diagnostiqueur. La

». Il paraît judicieux que le diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de démolition ou de réhabilitation significative de certains bâtiments indique bien les filières de recyclage existantes. Il s'agirait non seulement de responsabiliser plus encore les maîtres d'ouvrage, mais aussi d'éviter les erreurs dans le réemploi ou la valorisation desdits matériaux faute d'un recyclage satisfaisant. En outre, cela permettrait un gain de temps dans l'ensemble du processus. Rappelons que le diagnostic « déchets » est un enjeu important important pour l'économie circulaire, dans la mesure où, en 2014, le secteur du bâtiment et des travaux publics a produit 70 % des déchets totaux en France, soit 228 millions de tonnes. Il est donc essentiel de faire respecter cette obligation

réutilisable ». Cette précaution est fondamentale, en particulier pour des impératifs de santé publique. De plus, cette précision contribue à clarifier le rôle et les responsabilités qui incombent, d'une part, au maître d'ouvrage, et, d'autre part, à l'organisme qui réalise effectivement le diagnostic.

Nous souhaitons rendre public et librement consultable ce diagnostic, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce pourrait être consultable en mairie, en préfecture et/ou sur internet. L'objectif est bien évidemment de garantir est bien évidemment de garantir une meilleure information du public, notamment de permettre aux acteurs intéressés de se préparer à la gestion de ces déchets, assurant ainsi leur meilleure prise en charge au bénéfice de tous. Il s'agit d'en particulier d'avoir une information de l'ensemble du public sur des déchets pouvant entraîner des conséquences en matière de santé. Quel

un organisme agréé d'opérer un diagnostic des produits se situant dans l'immeuble à réhabiliter ou à démolir, est une très bonne chose. On demande aussi que ce diagnostic soit transmis à un organisme désigné par l'autorité administrative. Or je ne

d'un amendement rédactionnel.

satisfait par d'autres dispositions. Dans la législation actuelle, aucun dispositif n'est prévu pour récolter l'ensemble des diagnostics. Seules les informations qui viennent du recollement sont transmises à l'Ademe. En soi, cet article vient enrichir la récolte d'informations et renforcer la traçabilité. Comme le Gouvernement envisage que les diagnostics et les informations qui viennent du recollement soient transmis directement à l'Ademe pour s'assurer du respect de l'obligation réglementaire par les maîtres d'ouvrage et que l'Ademe est un établissement

Néanmoins, je considère que la réalisation d'un tel diagnostic, relatif à des produits, matériaux et déchets particuliers, nécessite de mobiliser des compétences qui soient reconnues. La question de la formation et de l'habilitation

Le projet de loi entend renforcer la qualité de ce diagnostic, actuellement très variable selon les chantiers, en prévoyant que les personnes chargées de l'établir présentent des garanties de compétence. Au regard de la technicité des informations et des enjeux de gestion de ces déchets, qui peuvent contenir des substances dangereuses, il conviendrait plutôt de faire référence à des critères de qualification.

dans le code de la construction et de l'habitation, par exemple pour garantir l'impartialité du contrôleur technique chargé de contrôler le fonctionnement des ascenseurs. Ainsi, ce contrôleur technique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à lui ni avec l'entreprise chargée des travaux ou de l'entretien. Par conséquent, pour prouver cette indépendance, il faudrait produire une attestation.

-, mais il n'existe pas aujourd'hui de moyen juridique permettant de faire la preuve du recyclage effectif des matériaux. Par ailleurs, les professionnels du recyclage ont besoin d'avoir accès à des informations sur l'origine des déchets qu'ils recyclent. Depuis 2014, au sein de la plateforme collaborative Démoclès, l'ensemble des parties prenantes concernées élabore divers outils, afin de faciliter le recyclage des déchets du bâtiment. Dans ce cadre, un modèle d'outil de traçabilité a été réalisé. Pour mettre en place celui-ci, il est maintenant nécessaire de le rendre obligatoire, afin de ne pas pénaliser les entreprises vertueuses qui pratiquent le recyclage, mais qui ne peuvent pas le démontrer, face à des entreprises concurrentes moins soucieuses de leur responsabilité environnementale. Le financement de cet outil par tous les acteurs permettra également de les impliquer et de garantir l'indépendance de la plateforme par rapport aux entreprises produisant des matériaux. De plus, les études de faisabilité des dispositifs de traçabilité montrent que le coût pour chacun des acteurs serait inférieur au coût d'une mauvaise gestion des déchets.

Pour ce faire, nous devons nous aider des dispositifs et des outils existants. D'après moi, le, ou bâti immobilier modélisé- BIM -, en fait partie. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, cet outil permet à l'ensemble des acteurs impliqués dans un projet de construction de partager leurs données tout au long de l'évolution du projet, depuis sa programmation jusqu'à son exploitation. Il permet également de modéliser les bâtiments existants, en y intégrant des éléments d'exploitation, voire de fin de vie, permet d'anticiper la déconstruction et de mettre en place une démarche d'économie circulaire. Il n'y a pas que le BIM ; le cahier numérique peut aussi être un outil. Cette proposition permet d'ouvrir la discussion. Cela devra se faire évidemment de manière échelonnée, mais nous devons fournir à nos professionnels du bâtiment tous les outils nécessaires pour arriver à nos objectifs en matière d'éco-conception.

Actuellement, lorsque les bâtiments nouveaux intègrent un taux minimal de matériaux biosourcés, c'est-à-dire issus de la biomasse végétale ou animale, et qu'ils répondent à certaines caractéristiques, ces bâtiments peuvent obtenir le label « Bâtiment biosourcé » ; c'est positif, mais largement insuffisant. En effet, d'après une étude du Gouvernement sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés, les matériaux biosourcés occupent seulement 6 % à 8 % des parts du marché de l'isolation rapportée ; c'est extrêmement peu.

L'effort que l'on doit produire sur les déchets du bâtiment, qui représentent un quart du volume global des déchets produits, passe prioritairement par une meilleure éco-conception des bâtiments, ce qui devrait nous conduire collectivement à poser la question de l'utilisation plus importante et systémique des matériaux biosourcés. Quel l'avis de la commission ? Il ne paraît pas réaliste de privilégier systématiquement, dans le cadre de la commande publique ou dans tout autre cadre, l'utilisation de matériaux biosourcés lors de la construction ou la rénovation de bâtiments.

du code de l'environnement dispose que la commande publique doit prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre des matériaux et le stockage du carbone au sein des matériaux de construction, ce que visent les matériaux biosourcés. La commande publique doit aussi veiller « au recours des matériaux issus de ressources renouvelables qui correspondent également aux matériaux biosourcés. Enfin, les professions du bâtiment bénéficient déjà d'une sensibilisation aux enjeux de la transition, dans le cadre du label «

de relocaliser l'emploi et de créer de nouvelles filières et elle favoriserait un développement économique s'articulant avec une économie sobre en émissions de carbone et en production de déchets. Le secteur du bâtiment est en effet l'un des secteurs les plus émissifs de gaz à effet de serre, beaucoup de mes collègues l'ont dit. De plus, l'utilisation du béton, qui a un fort impact environnemental, n'est pas neutre, notamment parce que sa fabrication exige l'importation de beaucoup de sable. Aujourd'hui, des solutions de remplacement existent ; elles sont le plus souvent préconisées par les architectes, qui, au-delà des plans de construction, formulent des indications sur les matériaux utilisés. Je pense, par exemple, au chanvre, mais également à la brique, ou encore à certains matériaux capables de retenir les gaz à effet de serre, autant d'atouts à valoriser la paille, le bois, notre pays n'en manque pas, et il ne manque pas non plus d'atouts pour la transition écologique. Nous souhaitons donc qu'un rapport recense l'ensemble de ces expériences et préconise les évolutions législatives favorisant l'utilisation de tels matériaux

La priorité des pouvoirs publics doit être la prévention de la production des déchets. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons globalement regretter sur ce projet de loi qui, au contraire, met l'accent sur la fin de vie des produits plutôt que sur leur réduction à la source. L'ensemble des acteurs de l'économie circulaire, notamment de l'économie sociale et solidaire, témoigne par ailleurs de la difficulté de mener des politiques opérationnelles, faute de financements à la hauteur. Il nous semble donc prioritaire d'axer les financements sur l'amont de la production de déchets, afin d'encourager la réduction des déchets à la source. L'essor de cette économie est essentiel d'un point de vue écologique, mais également parce qu'elle est potentiellement fortement génératrice d'emplois non délocalisables. Ces financements supplémentaires sont attendus pour, notamment, financer des initiatives locales et nationales de prolongement de la durée de vie des produits et de l'économie de la réparation, mais aussi pour identifier les activités qui ont besoin de soutien pour être rentables et pour se développer.

Il s'agit enfin d'accompagner les collectivités, qui souffrent de la baisse des dotations, dans la définition de leurs besoins de formation, et de conduire des programmes d'études et de recherche dans le domaine de la prévention. La question du financement reste bien la grande absente de ce texte. Pourtant, la prévention et le passage à une économie plus décarbonée exigent des financements nouveaux, et le Gouvernement doit s'engager, faute de quoi ce texte ne sera qu'une série de mesurettes à la portée limitée. Quel

Estrosi Sassone. La commande publique constitue un levier important pour déployer l'économie circulaire, notamment en matière de réemploi. Certains besoins peuvent être couverts grâce à cette solution, qu'il convient d'encourager. Toutefois, les besoins de la commande publique présentent de nombreuses spécificités, auxquelles les produits issus du réemploi ne peuvent pas toujours répondre : sécurité du matériel, notamment informatique, volume,

forcément. C'est notamment le cas en ce qui concerne les matériels de bureautique et les matériels médicaux par exemple. Il convient donc d'étudier avec attention les besoins en matière de réemploi, avant de se fixer des objectifs contraignants au titre de la commande publique. Aussi, l'amendement proposé vise à évaluer les besoins et le potentiel de réemploi associé à la commande publique.

constituait une étape indispensable à la transition vers une économie circulaire. La proposition 44 de la feuille de route prévoit notamment d'intégrer l'économie circulaire dans les stratégies de commandes publiques à travers la charte d'achat public durable ou encore l'abaissement du seuil à partir duquel le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables L'article 6 , introduit en commission, s'inscrit dans cette dynamique, que nous avons toutefois jugée un peu timide. Compte tenu de la nécessaire exemplarité de l'État et des collectivités et de la grande force de frappe économique de leurs stratégies d'achat, il nous paraît indispensable de préciser qu'un taux de 10 % de produits issus du réemploi est un minimum à atteindre.

Cet amendement vise à préciser que les produits réemployés doivent respecter les normes de sécurité et de qualité environnementale, afin d'éviter que des acteurs peu scrupuleux n'utilisent ce nouveau levier pour mettre sur le marché des produits qui ne respecteraient pas les critères de qualité et de sécurité s'imposant lors de la mise en marché, et cela au détriment du consommateur final. C'est un risque dont il est nécessaire de tenir compte, notamment pour les équipements électriques et électroniques, par exemple. Il s'agit non pas de vider de sa substance l'objectif d'encouragement du réemploi, mais d'introduire un garde-fou à l'égard de ceux qui pourraient profiter de ce levier pour mettre sur le marché des produits potentiellement dangereux pour le consommateur ou l'environnement.

un avis défavorable sur ces trois

Mme Maryse Carrère. Cet amendement vise à compléter les amendements précédents sur la commande publique, toujours dans un souci d'exemplarité des pouvoirs publics en matière d'économie circulaire. Les renouvellements de matériel sont fréquents dans l'administration et les collectivités locales. Nous souhaitons favoriser l'inscription de ces matériels dans le circuit du réemploi solidaire. Cet amendement a ainsi pour objet d'inciter l'État et les collectivités à signer des conventions avec des structures de l'économie sociale et solidaire, afin de multiplier les dons de biens qui sont en bon état et voués à être jetés.

impliquent de tout mettre en oeuvre pour créer des conventions de partenariat visant à faire primer une intelligence collective et participative de l'économie circulaire de proximité. C'est d'ores et déjà le cas dans de nombreuses agglomérations, dont Évreux Portes de Normandie, où je suis élue et où les ressourceries ressourceries et recycleries ont le droit de venir récupérer des déchets en déchetterie ou sur des points de collecte spécifiques, afin de les revaloriser, par la réparation ou la création de nouveaux objets à partir des matériaux. Les dispositions de cet amendement partent d'une vraie bonne idée, qui est d'associer les acteurs de l'économie sociale et solidaire à la collecte et au traitement des déchets ménagers dans les territoires,

pour les collectivités et l'État, de privilégier, dans le cahier des charges de leurs appels d'offres, évidemment à prix et à caractéristiques techniques équivalents, des produits issus du réemploi ou de recyclage, dans une proportion

issus du recyclage de déchets pouvant être utilisés en substitution de matières premières vierges. La réutilisation desdites matières premières est un bon moyen de lutter contre le productivisme délétère, qui participe à la raréfaction de nos ressources. Les bienfaits du recyclage sont aujourd'hui reconnus et prouvés scientifiquement. Celui-ci permet en effet d'éviter l'émission de 22,5 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 100 % des émissions du trafic aérien annuel, et d'économiser 123,5 térawattheures d'énergie par an, soit l'équivalent de 18 réacteurs nucléaires en France. Pour cette raison, l'État français a pris l'engagement de tendre vers 100 % de plastique recyclé et l'Union européenne vise l'incorporation de 10 millions de tonnes de matière plastique recyclée à l'horizon 2025. Cependant, la France n'arrivera pas à atteindre cet objectif si son droit reste inchangé. Le présent amendement tend donc à répondre à cette attente, en créant une obligation progressive d'incorporation de matières premières recyclées dans certains produits, afin de permettre leur mise sur le marché.

Il nous semble que fixer un pourcentage de réemploi pour chaque type de produit est très contraignant, donc trop rigide. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable

la fois la pérennité de cette technologie issue d'une recherche exclusivement française, le développement d'entreprises et le maintien d'un certain nombre d'activités. Je pense en particulier, en tant que Vendéen, à l'usine de pneumatiques pour poids lourds de La Roche-sur-Yon, dont les 680 salariés sont aujourd'hui sur la sellette.

inciter les collectivités et l'État à privilégier, dans leurs commandes publiques, les pneus rechapés plutôt que des pneus neufs, à prix et à qualité cette mesure accroîtra de manière significative les carnets de commandes d'un secteur en perte de compétitivité et menacé par la concurrence internationale. le secteur subit violemment l'importation de pneus venus d'Asie, de mauvaise qualité et à l'impact environnemental désastreux. Nous devons protéger les emplois industriels notamment ceux de l'usine Michelin à Avallon, dans l'Yonne, qui est la seule du groupe à faire du rechapage et dont les performances économiques sont aujourd'hui remises en question par la direction du groupe. de cette mesure de bon sens aura aussi un impact écologique positif et permettra un gain financier pour le pouvoir adjudicateur. Elle s'inscrit pleinement dans la logique de l'économie circulaire.

qui permettra de réduire nos dépenses, nos émissions de CO2 et notre dépendance aux matières premières et de créer de nombreux emplois non délocalisables. Parmi ces derniers, on trouve les emplois liés au rechapage des pneus, qui ont beaucoup souffert ces dernières années avec l'arrivée des pneus asiatiques low cost. L'État et les collectivités gèrent en propre plus de 41 000 poids lourds, ce qui représente 100 000 pneumatiques à changer chaque année, auxquels on peut ajouter toutes les flottes gérées par délégation de service public. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la nécessaire exemplarité de la commande publique. Les pouvoirs publics doivent utiliser ce levier pour favoriser, d'une part, une économie plus vertueuse et, d'autre part, n'ayons pas peur de le dire, les initiatives et les innovations françaises lorsqu'elles sont en adéquation avec l'objectif recherché. C'est entièrement le cas des pneus rechapés, qui réduisent de 70 % le besoin en matières premières et correspondent à 50 kilos de déchets en moins à recycler. Pour les finances de nos collectivités, c'est aussi un gain en termes de durée de vie, puisque celle-ci peut être doublée. À qualité égale, c'est même un gain direct, puisque le pneu rechapé coûte jusqu'à 40 % moins cher. Pour toutes ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, de voter en faveur de ces amendements.

scolaire. De nombreuses structures se sont emparées du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation. Toutefois, aucune évaluation n'a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournies et pour s'assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.

précise la place des producteurs dans la problématique de l'économie circulaire et de la limitation du gaspillage, je souhaite évoquer deux pistes qui n'ont pas été assez approfondies. Il s'agit tout d'abord de la lutte contre l'obsolescence programmée. Vous lui préférez la réparabilité, certes intéressante, mais pas suffisante. La loi de 2015 visait à sanctionner l'obsolescence programmée et à expérimenter, afin de mettre derrière ce concept plus d'effectivité. Il est en effet difficile de donner au consommateur une information claire et lisible sur la durée de vie des appareils, et donc d'empêcher le délit d'obsolescence programmée,

des marchés. Au final, il est essentiel de bien préparer l'organisation des filières, les process de production et de déterminer le taux d'incorporation de matières premières recyclées pour lesquelles les industriels devront utiliser des outils de traçabilité harmonisés à l'échelon européen leur permettant de connaître l'origine de la matière utilisée par leurs fournisseurs. Des contrôles devront par ailleurs être assurés par un organisme tiers-

La prise en compte du taux d'incorporation de matières recyclées dans les différents produits et matériaux est importante, mais elle ne peut être le seul critère pour certains matériaux. Je pense, par exemple, à l'aluminium l'augmentation du taux d'incorporation dans un produit peut se faire au détriment de son empreinte environnementale et carbone. Certains produits peuvent venir de loin, voire de très loin, et être conçus dans des conditions environnementales qui ne sont pas compatibles avec nos objectifs et nos standards français. L'amendement n° 429 rectifié, présenté

488 rectifié reprend en réalité plusieurs éléments déjà introduits en commission : prise en compte du bilan environnemental global dans la détermination de l'obligation d'incorporation de matière recyclée, décret définissant les règles de calcul du taux, contrôle afin de ne pas entraîner une situation de concurrence déloyale pour la production

je leur demande de bien vouloir le retirer. L'amendement n° 579 est pleinement satisfait par la modification introduite en commission qui vise à rappeler que l'obligation d'incorporation de matière recyclée n'est imposée que sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d'incorporation soit positif.

de matière recyclée, ce qui reviendrait à exclure la mise en place d'un taux minimal pour un certain nombre de matières.

imposée l'obligation d'incorporation de matière recyclée. J'espère que cette disposition permet de lever vos doutes et votre inquiétude. Enfin, je rappelle que la commission a adopté un amendement rappelant que l'obligation d'incorporation de matière recyclée n'est imposée que sous réserve

Cette disposition permet aussi de définir les taux d'incorporation réglementaires pour d'autres catégories de produits, afin de dynamiser la demande en matières recyclées.

À défaut, vous placez tout simplement l'industrie papetière française en situation de distorsion de concurrence négative. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays ; je maintiens donc mon amendement.

vote. Je demande quelques précisions. L'amendement tel qu'il est rédigé concerne tous les matériaux à l'exception de ceux qui sont issus des matières premières renouvelables.

prévues par le projet de loi. Nous pensons, de ce point de vue, qu'il est important de préciser que seront déterminés par décret les critères d'évaluation et les méthodes de calcul approuvées pour identifier et garantir l'origine de la matière.

le présent amendement vise à instaurer un objectif minimal de mise sur le marché de bouteilles réutilisables applicable aux plus grands metteurs sur le marché. de l'énergie -l'a montré, le système de consigne pour réemploi est très vertueux sur le plan environnemental, mais à la condition que son utilisation atteigne un certain seuil. C'est la massification des volumes d'emballages consignés et du maillage d'infrastructures correspondant qui permet d'optimiser le système. Cette solution est par ailleurs plébiscitée par la population, comme le montre également l'étude de l'Ademe, qui établit que les consommateurs sont prêts à adhérer à ce type de dispositif, que ce soit par conviction environnementale ou par intérêt économique, pour récupérer le montant de la consigne. Cette proposition vise donc à donner une orientation claire aux entreprises productrices de boisson pour les inciter à investir dans des solutions de réutilisation des emballages, des lignes de lavage ou des lieux de stockage. L'instauration d'un quota d'emballages réutilisables est une solution qui s'appuie sur l'existant, puisque la plupart de ces entreprises disposent déjà d'une ligne d'emballages réutilisables à destination des cafés, hôtels et restaurants, secteur des bouteilles et fûts sont toujours lavés avant d'être de nouveau remplis. On constate malgré tout, aujourd'hui, une tendance à la baisse de l'utilisation de ce système. Instaurer un quota de bouteilles réutilisables permettrait également d'enrayer cette tendance dans le secteur de la restauration et d'inciter les entreprises à préserver ces gammes réutilisables et à s'appuyer sur elles pour développer ce système la consigne. Une telle mesure est par ailleurs encouragée par la directive européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui donne la possibilité aux États de définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs et un pourcentage minimal d'emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d'emballages. Nous proposons, par cet amendement, que ce quota soit mis en place par décret, ce qui laisse la possibilité d'ouvrir une concertation avec les acteurs. En outre, la date de 2023 offre aux metteurs sur le marché un temps d'adaptation leur permettant de se conformer à cette réglementation. Il s'agit donc d'une mesure réaliste et nécessaire pour enfin limiter la production de déchets, la pollution et le gaspillage énergétique qui y sont associés.

Je ne suis pas favorable à ce que nous inscrivions dans la loi un objectif aussi précis pour les bouteilles, en tout cas pas sur le mode que vous proposez, mon cher collègue. Il me semble préférable de s'appuyer sur des incitations et sur les objectifs de réemploi qui vont être mis en place pour chaque filière, ainsi que dans les cahiers des charges, lesquels seront contrôlés

La refondation des filières REP prévue par le projet de loi crée par ailleurs un système de bonus-malus sur les éco-contributions, c'est-à-dire une modulation des éco-contributions en fonction de l'impact environnemental des emballages.